selon l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, un foyer qui s'attendait à payer 1 030 euros d'électricité pour l'année en janvier 2021 devra finalement s'acquitter d'une facture de 1 400 euros. Les 100 euros de chèque énergie ne suffiront pas, ni pour les plus pauvres ni pour tous les autres. d'une baisse substantielle du pouvoir d'achat, à laquelle s'ajoute la hausse continue, depuis plusieurs semaines, du prix des carburants. Pour autant, rien n'est prévu dans le projet de loi de finances pour faire contribuer les grands groupes pétroliers et les acteurs de l'énergie au financement et, ainsi, baisser réellement, pour tous nos concitoyens, le coût de l'énergie. Comptez-vous réellement ne pas mettre à contribution ces grands groupes pour l'effort de solidarité ?

rappelle l'augmentation de la prime d'activité, pour 4,4 millions de foyers, la suppression des cotisations chômage et maladie, pour 29 millions d'actifs, la baisse des impôts, notamment de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la revalorisation du traitement des professionnels de santé et des fonctionnaires les moins bien rémunérés. Voilà des actions concrètes,

au troisième trimestre ! Comme vous, nous avons écouté un président devenu candidat hier soi. Il n'a pratiquement pas abordé la première préoccupation des Français : le pouvoir d'achat. À l'inverse,

C'est pourtant de cela que les Français ont besoin ! En outre, les chèques préélectoraux ne compensent en rien la hausse de l'énergie et du carburant. Il y a urgence à offrir, dès à présent, aux aux Françaises et aux Français, les moyens de vivre dignement de leur travail. Il faut sortir de cette spirale qui plonge, jour après jour, de plus en plus de nos concitoyens dans la précarité. Ces femmes et ces hommes ne sont pas les coupables des difficultés de notre pays ; ils en sont aujourd'hui les premières victimes. La valeur travail ne se décrète pas, madame la ministre. Elle s'incarne, par l'ouverture immédiate de négociations pour la revalorisation du SMIC, des salaires et des pensions de retraite ! La parole est à M. Didier Rambaud, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Préserver la mission historique de service public attribuée à La Poste, malgré un déficit significatif lié à la baisse structurelle des volumes et aux conséquences de la crise sanitaire : l'État l'avait promis ; la promesse sera tenue Nos collègues Patrick Chaize, Pierre Louault et Rémi Cardon avaient estimé, dans leur rapport sénatorial, qu'une dotation budgétaire était nécessaire pour que La Poste continue à assurer un service postal universel sur tout le territoire. Cette dotation, mes chers collègues, nous l'avons nous l'avons ! Nous saluons le respect de cet engagement, madame la ministre. Le Gouvernement réaffirme son action en période de crise, avec deux priorités : soutenir notre économie et préserver les services publics de proximité, auxquels les Français sont attachés. Toutefois, des attentes, des interrogations, des inquiétudes demeurent. Elles sont nombreuses, parfois excessives, mais souvent légitimes. La peur du délitement et de l'éloignement des services publics est une réalité : nous ne pouvons la nier. Face à ces craintes, comment maintenir des services publics de proximité et de qualité dans notre pays, plus particulièrement dans les territoires ruraux ? Les attentes de nos concitoyens sont fortes. Nous devons poursuivre nos efforts pour répondre au sentiment d'abandon ou de déclassement, qui contribue à la crise de confiance entre les citoyens et les élus.

La parole est à M. Bernard Jomier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

pour protéger les Français. Aujourd'hui, nous faisons face à une recrudescence de l'épidémie. Ce n'est donc certainement pas le moment de se poser la question

Mais nous avons le sentiment que, avec ce passe sanitaire, vous êtes en train de changer de paradigme sur la question du contrôle. Car, de fait, vous étendez le recours à cet outil sans qu'on en perçoive bien les limites ; vous étendez le champ des contrôles systématiques, en lieu et place des contrôles aléatoires et, qui, dans une société démocratique et de liberté, sont les plus répandus. C'est là que se situe une interrogation profonde pour les parlementaires que nous sommes,

vouer. Cette année, la production de miel en France s'avère deux fois inférieure à celle de l'année dernière- la production se trouvait pourtant déjà en déclin. Les causes sont forcément multiples : météorologie, dérèglement climatique, emploi de pesticides. En dépit des immenses efforts de nos agriculteurs, viennent toutes participer à la perte de la richesse et de la biodiversité. Ce phénomène ne serait pas plus alarmant que les autres signaux de ce déclin si Albert Einstein n'avait pas prédit que la fin des abeilles, véritables indicateurs biologiques, annoncerait probablement la fin de l'humanité.

Cet observatoire est chargé de sélectionner des espèces d'abeilles plus résistantes, dans l'attente d'un environnement moins agressif pour elles, donc pour nous. Très prochainement, un arrêté Abeilles devrait paraître, au sujet duquel des désaccords relatifs à l'encadrement des heures d'autorisation d'épandage se font jour. met en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre une apiculture soucieuse et une agriculture vertueuse. Mais nous avons dû, dans la douleur,

le monde est face à son destin. La pandémie n'est pas terminée, faute d'avoir ouvert les brevets des vaccins et joué la solidarité mondiale ; le virus continue de circuler et de nous menacer. L'avenir de l'humanité, notre capacité à préserver une planète habitable pour l'espèce humaine, se joue en ce moment même à Glasgow. Dans ce contexte, alors que nous devons plus que jamais imaginer le monde solidaire et coopératif d'après, la France s'apprête à prendre la présidence de l'Union européenne. C'est le moment, légitime, que choisit le Président de la République pour s'adresser à la Nation : 27 minutes de discours ; 27 minutes pour dessiner non pas le monde de demain, mais le monde d'hier, voire d'avant-hier. Le travail invoqué comme un mantra, son corollaire de stigmatisation de toutes celles et tous ceux qui en sont exclus, la croissance, le productivisme, le nucléaire tous ces étendards des Trente Glorieuses sonnent si faux dans la bouche d'un homme qui n'a connu que la crise structurelle d'un capitalisme incompatible avec la préservation du vivant et la justice sociale. de la République est sidérant : sur l'investissement en faveur de la santé, quand l'hôpital a perdu 5 700 lits au milieu de la pandémie ; comme sur la pauvreté, alors que la misère s'intensifie toujours. Face au concours Lépine des mesures ineptes et injustes proposées par les candidats LR lundi soir sur LCI, Emmanuel Macron est venu rappeler à tous ceux qui voudraient l'oublier que la droite, c'est lui

concitoyens de s'élever par le travail, d'obtenir un meilleur salaire et une meilleure place dans la société. Oui, il faut faire entrer en vigueur la réforme de l'assurance chômage. Oui, il faut que Pôle emploi multiplie les actions en direction des entreprises et des demandeurs d'emploi, y compris les contrôles-

ministre, vous êtes satisfait ! Pourtant, on ne construira pas l'avenir avec les lunettes du passé ; on ne luttera pas contre le dérèglement climatique sans changer de modèle ; on ne réduira pas les inégalités en s'acharnant sur les plus démunis. Notre avenir sera écologique et solidaire ou ne sera pas

Pour l'heure, leur mission consiste essentiellement à définir les critères d'attribution des subventions. Les décisions concernant les nouveaux projets seront rendues en début d'année prochaine, en janvier ou en février selon les cas, pour un versement effectif en mars 2022. Nous le savons tous ici, il s'agit d'un moment important pour les collectivités territoriales et les élus locaux. L'attribution de la DETR a de puissants effets d'entraînement pour le tissu des entreprises situées dans les départements ruraux. Chaque année, les procédures d'attribution sont suivies de près par les élus. Mais cette année, le contexte économique devrait donner une tournure un peu particulière à ces rendez-vous. Et pour cause, l'inflation fait son grand retour. Nous en connaissons les raisons macroéconomiques : compte tenu de la forte reprise en sortie de crise, la demande est importante et la pression s'accroît sur les matières premières et l'énergie. De façon très concrète, cela se traduit par une augmentation très forte des coûts des projets. Les hypothèses sur lesquelles les dossiers ont été bâtis, préparés de longue date par les porteurs de projets, sont devenues caduques. Et les plans de financement risquent fortement de déraper. Dans ce contexte, madame la ministre, ma question est assez simple : alors que le Sénat examinera tout prochainement le projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement envisage-t-il de réviser l'enveloppe globale de la DETR pour prendre en compte les effets de l'inflation ? Plus généralement, et au-delà de ce dispositif particulier, quelles sont les réponses que le Gouvernement peut apporter aux élus locaux, qui craignent de voir les budgets prévisionnels déraper à cause de l'inflation ?

un plaisir de vous répondre. Je partage votre préoccupation concernant les conséquences de l'inflation sur les coûts des travaux publics. C'est un sujet qui concerne en premier chef les collectivités, lesquelles réalisent la majeure partie de l'investissement civil. quelques éléments de contexte : la hausse des prix a été mesurée en 2020 à 0,5 %. Elle redémarre en 2021 et 2022, tirée par la hausse des prix de l'énergie. Cependant, cette hausse ne se répercute pas forcément sur tous les chantiers. Souvent, le coût final correspond au devis signé entre les maîtres d'ouvrage et l'entreprise. D'ailleurs, les remontées des collectivités locales sur ce sujet

Je pense notamment aux impôts assis sur la base locative cadastrale, revalorisés chaque année en tenant compte de l'indice des prix. Le taux d'actualisation pour l'année 2022 n'est pas encore connu, car il dépend des données de novembre 2021. Je pense aussi à la TVA, qui dépend du prix des consommations. En 2022, la hausse du produit de la TVA pourra être de 5,8 % et rapporter 400 millions d'euros aux intercommunalités, 800 millions d'euros aux départements et la même somme aux régions. Bien entendu, nous continuerons à regarder la situation des collectivités de près. Le Gouvernement soutiendra les collectivités, comme il l'a toujours fait depuis 2017, et surtout en ces temps très troublés.

Monsieur le Premier ministre, présent il y a quelques jours à l'Élysée, j'ai été ravi d'y entendre le Président de la République appeler, dans le cadre du plan France 2030, à un élan de réindustrialisation. Mais de la parole aux actes il y a parfois un fossé, comme le cas suivant l'illustre concrètement. En Meurthe-et-Moselle, à Pont-à-Mousson, Saint-Gobain, fleuron de l'industrie française en matière de tuyaux d'eau en fonte ductile, qui emploie 2 000 personnes, qui est

réciprocité normative, puisque l'Inde est un pays entièrement fermé aux exportations. Monsieur le Premier ministre, confirmez-vous cette information, la justifiez-vous ? Surtout, quelle est votre stratégie pour parvenir à la nécessaire réindustrialisation de la France ?

Vigilants sur le projet industriel, qui aurait pu changer la trajectoire de ce site, pour nous assurer que ce dernier ne tombe pas entre des mains peu favorables d'un point de vue industriel. Vigilants pour rendre plus aisées et automatiques les clauses sociales et environnementales aux acheteurs publics locaux, qui leur permettent de mieux prendre en compte la valeur extrafinancière des conduites en fonte vendues par Pont-à-Mousson. Vigilants donc, en changeant la loi pour cela. Vigilants en validant un soutien au titre du plan de relance de 2,5 millions d'euros pour l'installation d'un four électrique à Pont-à-Mousson, qui sera le plus grand d'Europe. Cette aide s'ajoute à l'ensemble de celles dont bénéficie Saint-Gobain au titre du plan de relance industriel, soit 10 millions d'euros au total. Dans le cadre de la rénovation thermique, on peut d'ailleurs penser que Saint-Gobain est l'un des principaux bénéficiaires du plan de relance. Croyez bien que nous sommes

et dont les conduites sont achetées par des collectivités locales, cherchent aujourd'hui à s'implanter eu Europe. De quoi est-il question ? D'avoir une entreprise qui produit en France avec des salariés français, dans des conditions de travail, des

mais : restructuration, fermeture d'un site. Le marché français est en surcapacité de 50 %. Comment voulez-vous nous faire comprendre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, un sondage de la revue vient de révéler que huit Français sur dix sont inquiets du niveau de la dette publique. Cantonner la dette covid ne suffit pas à la rembourser. Je souhaite donc savoir quelle est votre stratégie de désendettement. Hier soir, le Président de la République s'est félicité d'avoir géré la crise sanitaire en « maîtrisant notre déficit public ». Il a ajouté que ce déficit serait de moins de 5 % du PIB cette année. Or nous en étions restés à une prévision de 8,1 % du PIB. Disposeriez-vous d'éléments que nous ignorons pour l'étude du projet de loi de finances pour 2022 ? Dans ce cas, le Parlement pourrait-il en être destinataire, au lieu de débattre de chiffres obsolètes ? Madame la ministre, Les dépenses pour faire face à la crise sanitaire étaient nécessaires et nous les avons votées, en cautionnant ainsi l'endettement généré.

Mais le PLF 2022 est-il lucide ? Où est la trajectoire vertueuse que nous devons à nos créanciers ? Y a-t-il des chiffres que nous ne connaissons pas ? La France connaît-elle le secret de l'argent magique ?

et nous visons 5 % de déficit public en 2022. Il n'y a pas de magie dans ces chiffres, ils sont publics, nous les partageons avec vous, et vous allez être amenés à vous prononcer. Concernant la trajectoire dans la durée, vous savez que 165 milliards

ailleurs le FMI vient d'exhorter la France à faire des efforts, et je crois qu'il a bien raison. Si les taux d'intérêt remontent, la charge de la dette sera colossale. Il s'agit donc d'établir des budgets vertueux,

Ma question s'adressait à monsieur le Premier ministre et je remercie M. le ministre de la santé de me répondre, même si le sujet me semble un peu éloigné de ses préoccupations. Peut-être se sentira-t-il concerné ... En effet, monsieur le ministre, les jours passent et se ressemblent. Chaque jour, les annonces tombent, les millions et milliards se succèdent, si bien qu'il faut désormais une double page pour tout additionner : +30 milliards pour le plan d'investissement, +2 milliards pour le contrat d'engagement jeune, +4 milliards pour l'indemnité inflation, +2 milliards pour renflouer France Compétences ... Bref, en moins de trois

Chaque jour, ont lieu des États généraux. On travaille ! Les plus récents portent sur la justice, alors même que six textes ont été portés par votre gouvernement et par le précédent sur ce thème. Monsieur le ministre, je pourrais être plus longue, mais je n'ai finalement qu'une seule question : est-il moral de faire campagne avec l'argent des Français, en creusant la dette ?

Président de la République hier. Alors que nous attendions un discours sur la covid, nous avons finalement assisté à un discours de campagne présidentielle. Chaque jour, chaque soir, Emmanuel Macron achète son élection La parole est à Mme Catherine Conconne, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alors, attention ! Toutes les révoltes sociales dans la dite outre-mer, notamment celle de 2009, sont nées de la hausse des prix de l'énergie. Je vous appelle donc à agir dès maintenant, à ne pas attendre l'explosion. Je suis consciente que l'angle d'attaque ne saurait être la fiscalité. Les taxes État sont nulles, celles des collectivités plus que raisonnables. Côté brut, on connaît les conditions du marché. J'aimerais cependant attirer votre attention sur d'autres composantes de la fixation des prix, qui semblent manquer totalement de transparence. Arrêtons-nous un instant sur l'exemple très emblématique du gaz utilisé par de nombreux foyers - plus de 10 000 tonnes ont été consommées l'an dernier l'an dernier sur notre île. En deux ans, le prix du bidon a augmenté de 50 % ! Sur un montant de 32 euros, la moitié, soit 16 euros, représente des coûts de distribution. Si la part du transport et du revendeur de ce produit semble légitime - elle s'élève à un peu plus de 4 euros -, comment se décomposent les 12 euros restants sur les 32 du prix global ? Qui rémunèrent-ils, et sur quelle base ? On l'ignore, ou on en sait si peu ! Il y a une urgence de transparence. Il existe un sentiment d'injustice, qualifié de « pwofitasyon » en créole, qui perdure. Non, nos populations ne peuvent pas être toujours plus pauvres et payer toujours plus cher. Ce n'est pas acceptable ! Oui, il y a le chèque énergie. C'est un soulagement ponctuel, mais ce n'est pas la solution Madame la ministre, êtes-vous prête à lancer courageusement cette nécessaire mission transparence très attendue, afin de soulager les Ultramarins face à la flambée des prix ? L'État est-il prêt à enfin faire la transparence sur ces rémunérations d'intermédiaires et ces marges qui semblent frappées d'opacité

Cette indemnité concernera environ 38 millions de nos concitoyens, qui touchent moins de 2 000 euros net par mois, et près d'un million d'Ultramarins en seront destinataires. Tous seront concernés : ceux qui travaillent, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, les retraités ou les bénéficiaires des minima sociaux. Ces mesures sont des mesures de justice sociale et de lutte contre la précarité énergétique. Bien entendu, nous veillons à ce que l'application stricte de la formule de calcul des prix réglementés des carburants empêche toute marge indue.

qui bénéficiera également aux entreprises. Il y a donc une totale transparence. Les tarifs réglementés de vente du gaz de ville sont aussi gelés jusqu'à la fin de l'année 2022. Le coût de ce bouclier tarifaire ... Il faut conclure ! ... est de 5 milliards d'euros, le chèque énergie représente 600 millions d'euros, la prime inflation, 3,8 milliards

Monsieur le ministre des solidarités et de la santé, alors que le Gouvernement a prétendu piloter la crise sanitaire en fonction du risque de saturation hospitalière, il peut sembler surprenant que des lits soient massivement fermés à l'hôpital public.

En réalité, le manque de personnel oblige à laisser inoccupés bien plus que 6 % des lits. Dans les faits, ces lits sont bien fermés, mais seuls les lits fermés administrativement sont comptabilisés dans les chiffres officiels. À côté de cela, l'absentéisme et les démissions des professionnels de santé à l'hôpital augmentent sérieusement en raison de la dégradation progressive des conditions de travail.

? Pourquoi maintenir ces primes liées aux réductions de la masse salariale et des capacités hospitalières ? Madame la sénatrice Lassarade, je ne sais que vous répondre. Vous parlez de discordance entre des chiffres et énoncez, excusez-moi de vous le dire, des contre-vérités. Vous faites un amalgame, qui me paraît probablement lié à une mauvaise information : je me permets de le dire,

universitaires). Que nous dit-elle ? D'abord, qu'il y a plus de soignants dans les hôpitaux à l'automne 2021 qu'à l'automne 2019. Nous recrutons du personnel. Ensuite, elle nous dit que, sur

la France est un grand pays maritime et nous avons intérêt à préserver le potentiel qui en découle. Nous pensions que les accords liés à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe avaient été bien négociés, mais nous constatons, hélas,

Aujourd'hui, le problème est que cet accord n'est pas respecté. Nous ne pouvons pas faire des compromis au-delà de ce qui a été négocié, signé et ratifié par les parlements européen et britannique ces derniers mois. mois. Depuis dix mois, avec Annick Girardin, sous l'autorité du Premier ministre, nous travaillons avec l'ensemble des élus des régions concernées, les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne, et surtout avec les professionnels, pour obtenir ces licences de pêche. Nous les avons obtenues intégralement pour la zone économique exclusive,

il y a quelques jours, que nous étions prêts à prendre des mesures. Cette fermeté supplémentaire a amené à une nouvelle phase de dialogue avec les Britanniques. J'ai reçu la semaine dernière Lord Frost, qui s'occupe des négociations sur le Brexit, et je lui ai de nouveau parlé hier. Aujourd'hui même a lieu une discussion portant sur les deux points qui posent le plus de problèmes

face à ces difficultés temporaires concernant le mareyage et des activités de pêche. Nous mobiliserons toutes les sommes nécessaires. Mais ce que veulent nos pêcheurs, c'est surtout reprendre leur activité économique, et c'est cela que nous leur devons. nous partageons l'objectif que les patrons pêcheurs puissent rapidement reprendre leur travail. Cela fait onze mois que cette situation dure : il est temps que des solutions soient apportées. La France a voulu faire preuve de fermeté

et plus s'éloigne la perspective d'obtenir des solutions positives pour nos marins pêcheurs. Les inquiétudes ne cessent de monter sur les quais et il est important que des solutions soient amenées. Puisque les Assises de la pêche et des produits de la mer vont se tenir à Saint-Paul-de-Léon

financement de la sécurité sociale), nous sommes nombreux sur toutes ces travées à vous alerter et à faire des propositions en matière de lutte active contre les déserts médicaux. La loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé de 2019 a notamment prévu, à la demande du Sénat,

Le Gouvernement n'a pas mis en oeuvre cette disposition, alors qu'il s'y était engagé. Pourquoi ? Depuis, le nombre de nos concitoyens qui n'ont plus accès aux soins ne cesse de croître. Ils seraient désormais, selon la direction de la recherche, des La Cour des comptes le préconise, les maires le réclament, les familles l'exigent, les patients en ont besoin et notre responsabilité politique l'appelle : nous devons aller au-delà des mesures incitatives, qui ont leur sens mais qui ne suffisent pas, ne suffisent plus. Dans l'attente des effets du desserrement du, qu'il faut amplifier, nous devons donc

Désormais, même les professionnels de santé réclament des mesures plus fortes : conventionnement sélectif, stage post-doctorat ou encore zones franches médicales. Aussi, que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens ? La parole

que nombre de sénateurs ici présents, pourtant très sensibles, je le sais, à la cause des déserts médicaux, déposent des amendements tendant à supprimer toute disposition permettant de favoriser les coopérations interprofessionnelles et de rendre ainsi les Français moins dépendants à l'accès direct au médecin lorsqu'il n'y a pas de praticiens dans les territoires concernés.

Monsieur le ministre, la pénurie est peut-être globale, mais la responsabilité d'aujourd'hui est d'agir. Une loi a été adoptée en 2019, mais elle n'est pas appliquée. D'autres mesures doivent être mises en place, faute de quoi il y aura un réel problème d'accès aux soins pour nos concitoyens et la responsabilité en reviendra au gouvernement d'aujourd'hui. La parole

Par conséquent, quand ces aides ne sont pas versées à la date prévue, les agriculteurs doivent négocier des emprunts auprès des banques pour combler leur besoin de trésorerie. C'est justement le cas au moment où je parle,

! Monsieur le ministre, mes chers collègues, doit-on incriminer l'Europe pour ces retards, comme on a si souvent tendance à le faire, parfois à raison ? Dans ce cas d'espèce, ce n'est pas Bruxelles qui est en cause : l'argent est bien disponible, mais, pour qu'il soit versé aux agriculteurs, il faut que l'État français ait contrôlé l'exploitation S'agissant d'argent public, personne ici ne remet en cause la légitimité de ces contrôles, qui permettent de vérifier la conformité des productions agricoles. Ce que je déplore et qui est inadmissible, c'est que l'administration française n'ait pas les moyens d'effectuer ces contrôles dans les délais requis pour que les agriculteurs reçoivent les aides nécessaires à leur survie aux dates que vous aviez annoncées, monsieur le ministre. Par conséquent, qu'allez-vous faire pour que nos agriculteurs reçoivent leur prime le plus rapidement possible ? La parole

La parole est à Mme Laure Darcos, pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le ministre, l'hôpital public va mal et les soignants sont au bord de la crise de nerfs. Quand le Gouvernement communique sur les milliards d'euros mobilisés dans le cadre du Ségur de la santé, sur le terrain, les services peinent à assurer leurs missions auprès des patients. Remise en cause des vocations, multiplication des burn-out, pénurie de soignants, difficultés de recrutement ou encore fermetures de lit : l'hôpital fait face à des difficultés sans fin, dans le prolongement de la crise de la covid-19. Puisque vous avez dit à ma collègue Florence Lassarade qu'elle faisait des amalgames, je vais vous donner un exemple précis, des services de pédiatrie, qui sont dans une situation de tension extrême. Ces services doivent aujourd'hui traiter les conséquences de l'épidémie sur la santé des adolescents, dans un contexte de saturation totale des structures régionales Ils doivent aussi composer avec un départ massif des pédiatres vers le secteur privé, où ces professionnels échappent aux contraintes toujours plus lourdes de la permanence des soins. À titre d'exemple, le service de pédiatrie de l'hôpital d'Orsay, dans mon département, l'Essonne, a perdu quatre de ses six pédiatres, ce qui a conduit à la fermeture de douze lits, qui manquent désormais cruellement. La pénurie de personnel non médical, quant à elle, entraîne le gel de lits de pédiatrie et de néonatalogie dans tous les hôpitaux comme, par exemple, à Longjumeau. Enfin, pour ajouter à cette situation désespérante, la survenue précoce de l'épidémie de bronchiolite engendre un nombre record de consultations dans les services hospitaliers. Dans ce contexte se pose la question cruciale de la compensation de l'extrême pénibilité des gardes de nuit pour les médecins, qui s'élève actuellement à moins de 18 euros brut par heure. Nous savons que cette pénibilité se traduit par des départs multiples de l'hôpital public, en particulier dans les secteurs ne bénéficiant pas d'un calcul horaire du temps de travail des médecins, comme la pédiatrie et la gynécologie-obstétrique. Il s'agit d'un angle mort du Ségur. Monsieur le ministre, vous avez vous-même reconnu la situation de tension dans les services d'urgence, de pédiatrie et dans les maternités, lors de votre présence au salon de la Fédération hospitalière de France. Comptez-vous prendre une initiative forte en la matière pour éviter la catastrophe annoncée ?

Ensuite, il y a une charge de travail importante en pédiatrie, liée à l'activité de pédopsychiatrie que vous avez soulignée. Cette croissance de l'activité pédopsychiatrique, nous avions commencé de la constater avant la crise de elle se poursuit, voire s'accentue. De fait, jusqu'à 30 % des lits de pédiatrie générale sont occupés par des enfants qui relèvent de pédopsychiatrie. Nous avons en effet une véritable pénurie médicale en pédopsychiatrie et, là encore, nous sommes déterminés à en former bien davantage dans les années à venir.

les services d'urgence fonctionnent tant bien que mal, mais certains sont tout de même amenés à fermer. La pénurie d'urgentistes est telle qu'un système mercantile s'est mis en place, siphonnant les moyens financiers des hôpitaux et compromettant la prise en charge des patients.

Les élus sont prêts à toutes les compromissions pour chiper le praticien de leur voisin. Néanmoins, ce marché est malsain et les surenchères financières ne règlent rien, bien au contraire ; c'est d'ailleurs ce que l'on constate aujourd'hui. Depuis plus de dix ans, on nous dit chaque année qu'il suffit d'attendre un peu pour que les choses s'arrangent, mais c'est de pis en pis. Aussi ma question est-elle simple, monsieur le ministre : quand ?

? Vous avez évoqué le, mais, vous le savez bien, c'est en termes de temps médical qu'il faut raisonner ; je voudrais être certaine que les modélisations de vos services intègrent les changements de mode d'exercice, le salariat, la féminisation de la profession, le nombre de médecins et d'étudiants qui

tragédies est, hélas, longue. Ils sont arrivés au péril de leur vie en France ; ils y trouvent la mort plutôt que l'accueil. Ils veulent gagner la Grande-Bretagne pour s'y construire un avenir plus décent ; on les en empêche et, en attendant, ils errent dans les rues de Calais. Le prêtre Philippe Demeestère a fait vingt-cinq jours de grève de la faim ; deux autres personnes- Ludovic Holbein et Anaïs Vogel -l'ont accompagné dans cette action et poursuivent leur grève, afin de dénoncer la situation des quelque 1 500 migrants

rien de nouveau, rien de concret n'est sorti de ces négociations. Migrants et associations, eux, attendent un moratoire sur les évacuations pour l'hiver. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre de l'intérieur ? font-ils partie de votre vocabulaire ? La République a-t-elle, oui ou non, un devoir de fraternité à l'égard de gens, qui, avant d'être des clandestins, sont nos semblables, des humains ?

... Écoutez, on ne peut pas parler, le débat n'est pas possible. Je le regrette. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.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

dernière, nous avons adopté, en loi de financement de la sécurité sociale, une réforme majeure de l'accès précoce. Cette réforme, qui a profondément revu les mécanismes de prise en charge dérogatoire, a rénové le cadre de l'accès des patients à l'innovation, et ce même très en amont d'une autorisation de mise sur le marché

sans condition de gravité de la pathologie ni d'urgence. Il pourra, en outre, être ouvert à des spécialités présentant un service médical rendu important, mais avec une amélioration, même mineure, du service médical rendu, de I à IV.

Il ne faut pas que cette expérimentation conduise à bouleverser la réforme de l'accès précoce, mise en oeuvre depuis juillet dernier seulement, et dont tous les acteurs se félicitent. Derrière ces dispositifs, il y a des patients qui attendent : ne risquons pas de retarder l'accès des patients atteints de pathologies graves à des médicaments innovants. avons mis en place l'accès précoce : un médicament peut être autorisé, avant l'AMM, pour des maladies graves, rares ou invalidantes et sans autre alternative thérapeutique.

L'accès précoce et l'accès compassionnel ne sont applicables que depuis le 1 juillet dernier. Comment le Gouvernement peut-il déjà évaluer que ces deux modalités de mise à disposition de médicaments innovants sont insuffisantes pour « garantir un accès et une prise en charge immédiats des patients

En les empilant de nouveau et en déstabilisant le système chaque année, le Gouvernement va à rebours de son objectif. La critique d'une complexité due à de multiples modifications incrémentales, utilisée pour justifier la réforme de l'an passé, peut tout à fait s'appliquer, cette année, à celle de Enfin, l'inquiétude et les incertitudes soulevées par cette nouvelle expérimentation résident dans le fait que cet article dépasse les restrictions posées dans loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, puisqu'il autorise l'accès au marché et le remboursement de médicaments venant soigner des maladies qui ne sont pas rares ou graves et de médicaments n'étant pas évalués comme innovants, contrairement aux exigences

une réponse à d'autres besoins. Il y a bien un sujet concernant l'articulation avec la réforme des ATU, que nous avons votée l'an dernier, mais cela ne justifie pas la suppression de l'article.

Rien ne justifie cette restriction : l'alinéa 4, que je vous propose de supprimer, réserve le bénéfice de l'accès direct à une mise à disposition des patients, après l'évaluation de la Haute Autorité de santé, aux seuls médicaments n'ayant pu bénéficier de l'accès précoce tout en y étant éligibles.

Toutefois, en raison de la lourdeur de la procédure tant pour les agences que pour les laboratoires, le Gouvernement envisage de mettre en place une grille de remise augmentée pour l'accès direct par rapport à celle de l'accès précoce, et ce afin

Un amendement gouvernemental, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, a précisé que l'accès direct s'appliquait aux traitements innovants n'ayant pas obtenu au préalable une autorisation d'accès précoce. Cependant, le délai imposé aux industriels pour effectuer cette demande d'accès précoce apparaît peu réaliste et risque de rendre l'accès direct inopérant. En effet, les laboratoires pharmaceutiques, et à plus forte raison les petites entreprises et start-up, ne seront pas en mesure de déposer un dossier de demande d'accès précoce en France avant même la demande d'autorisation de mise sur le marché, surtout lorsqu'il s'agit d'une procédure centralisée européenne- les AMM européennes sont parfois délivrées près de deux ans après le dépôt de la demande. À ce stade, dans la grande majorité des cas, les entreprises ne disposent pas encore d'une vision suffisamment fine pour leur permettre de savoir si le traitement peut répondre aux exigences du dispositif d'accès précoce. Il convient donc de lever

elle-même présentés ? En tant que rapporteure, il me revient de conseiller le Sénat et de lui proposer une position cohérente en vue d'assurer la solidité du dispositif.

Partant du principe que l'essentiel des médicaments concernés par l'accès direct ne devrait pas être éligible à l'accès précoce, il ne nous paraît pas opportun- ce serait même contre-productif -de prévoir le dépôt systématique d'une demande d'accès précoce comme condition nécessaire. Par ailleurs, une question de cohérence des calendriers se pose avec une date butoir fixée à la date de demande d'autorisation de mise sur le marché qui ne semble pas en adéquation avec le fonctionnement réel des industriels et des autorités sanitaires.

sont infondées ? Il faut certainement faire confiance aux industriels et le Gouvernement veillera, par l'incitation des barèmes tarifaires à l'attractivité de l'accès précoce vis-à-vis de l'accès direct- croisons les doigts ! La solution de la commission n'est peut-être pas parfaite, monsieur le ministre, mais nous avons l'humilité de le reconnaître. Nous étions ouverts à la discussion, prêts à l'affiner. C'est la raison d'être du débat parlementaire. Face à une fin de non-recevoir et au dépôt de ces amendements, je ne suis pas dupe : la négociation sur cet article

Alors que le dispositif tend à permettre un accès rapide à l'innovation, il est important de garantir une rapidité de publication des actes réglementaires nécessaires. Le présent amendement vise donc à prévoir un délai maximum concernant l'arrêté de prise en charge.

Annie Delmont-Koropoulis. Cet amendement vise à supprimer la faculté qu'a le CEPS de fixer unilatéralement le prix d'un produit bénéficiant de l'accès direct, faute d'accord avec l'exploitant au bout de douze mois. Cette disposition a été introduite par amendement gouvernemental en séance Néanmoins, elle contribuerait à biaiser la négociation de prix. Le CEPS a désormais intérêt à ne pas arriver à un accord sur le prix, puisqu'il prendra la décision finale. Par ailleurs, c'est extrêmement dissuasif pour l'entreprise, qui pourrait se voir imposer unilatéralement un prix. Une telle mesure, qui possède donc un caractère désincitatif pour les entreprises, risque de rendre le dispositif inopérant. Faute d'accord sur le prix, il semble préférable de conserver l'accord-cadre négocié

en cas d'inscription au remboursement à l'issue de l'accès direct, de fixation du prix de manière unilatérale par le CEPS, faute d'accord dans un délai de dix mois. Il ne semble pas pertinent de revenir sur ce dispositif subsidiaire, qui préserve tout de même la durée des négociations avec le CEPS. La commission est donc défavorable

Or, selon une étude, entre 2007 et 2017, 268 médicaments ont été autorisés sur l'avis de l'Agence européenne des médicament, dont 39 au terme d'une procédure accélérée. Seuls 31 % de ces médicaments avaient une valeur thérapeutique élevée. Dans ce contexte, la mise en oeuvre d'un tel mécanisme pourrait contribuer à ce que la sécurité sociale solvabilise des médicaments qui n'amélioreraient pas réellement le service rendu. C'est un point auquel nous sommes, je crois, toutes et tous attachés. cet amendement, il s'agit donc de préciser à l'article 36 que l'évaluation intègre la dimension du service médical rendu. En effet, il convient que les procédures visant à réduire les délais de mise sur le marché des produits de santé

la porte à des abus, notamment en matière de prix, par un certain nombre de laboratoires. Toutefois, à partir du moment où Mme la rapporteure me dit que notre amendement prête à confusion et va à l'encontre de notre souhait, je le retire.

Afin de favoriser l'émergence, l'adoption et l'utilisation précoce d'innovations pionnières, il est ainsi proposé la mise en place d'un budget, décentralisé et dédié aux équipes pionnières. Ce budget serait serait strictement fléché vers des équipes hospitalières pionnières de centres de référence, et octroyé en contrepartie d'une collecte et du partage des données préliminaires quant à l'utilisation du dispositif médical innovant et de l'acte qui y est associé. L'accès à un dispositif médical innovant pour un patient et un professionnel de santé est théoriquement possible dès que le marquage CE est obtenu. Mais sa prise en charge par l'assurance maladie n'intervient

D'autre part, les méthodologies d'évaluation sont difficiles à satisfaire à un stade d'usage précoce d'un dispositif. La trop forte centralisation et le contrôle de l'accès aux budgets limitent par ailleurs fortement la rapidité d'accès au financement et freinent considérablement l'émergence de nouveaux usages positifs des innovations. De même, il est également très complexe pour un établissement hospitalier et ses équipes pionnières de financer de manière ces innovations pour permettre leur usage. Ces constats traduisent l'absence, aujourd'hui, en France,

? Cet amendement vise à permettre un nouveau circuit de financement de l'innovation, par le biais des dotations dédiées aux missions d'intérêt général (MIG). Une telle

Ensuite, les crédits MIG sont limités et permettent d'assurer de nombreuses missions, notamment d'enseignement et de recherche, mais aussi de vigilance et de veille épidémiologique : veille sanitaire, prévention et gestion des risques, intervention d'équipes pluridisciplinaires et coordination pour certaines pathologies spécifiques.

Elle est accompagnée par nos collègues Mathieu Darnaud, président du groupe d'amitié France-Asie du Sud-Est, et Jérôme Durain, président délégué pour le Bangladesh. Son Excellence Sheikh Hasina est en visite en France pour participer au Forum de la Paix, qui se tiendra à la fin de cette semaine à Paris. Elle échangera cet après-midi avec les sénateurs membres du groupe d'amitié France-Asie du Sud-Est. Le Sénat entretient d'excellentes relations avec le Bangladesh et avec le Parlement bangladais en particulier. Une délégation du groupe d'amitié s'y est rendue en 2019. Nos collègues avaient été reçus par la présidente du Parlement et le ministre des affaires étrangères, Son Excellence AK Momen, que nous avons accueilli au Sénat la même année pour un Forum économique France-Bangladesh. Le Bangladesh fête cette année le cinquantième anniversaire de son indépendance, mais aussi le centenaire de la naissance du « Père de la Nation, Bangabandhu », père de la Première ministre. Les relations entre la France et le Bangladesh sont anciennes ; elles se sont intensifiées récemment avec, en particulier, le développement de coopérations dans le domaine de la défense et de la lutte contre le terrorisme. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à Mme la Première ministre et à sa délégation la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour.

de créer une enveloppe consacrée à la prise en charge des actes de médecine génomique. La commission alerte depuis plusieurs années sur la nécessité de réviser le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN), afin de prévoir une meilleure prise en charge de certains actes comme les tests compagnons. Toutefois, conformément à la position habituelle de la commission sur les demandes de rapport, il s'agit, par cet amendement, de supprimer l'article.

Comment demander au Parlement d'abroger des dispositions, pour les rétablir deux ans après, sans étayer davantage sa motivation ? Si les échanges informels que j'ai pu avoir avec l'ANSM sont tout à fait rassurants sur les positions de l'agence et l'encadrement du dispositif et nous permettent de voter cet article,

n° 53 rectifié. Depuis l'arrivée du premier biosimilaire sur le marché français en 2006, le recours à ces médicaments, équivalents aux médicaments biologiques, mais, en moyenne, 30 % moins chers que leurs médicaments de référence, reste limité. Si la pénétration des biosimilaires à l'hôpital est estimée à 69 % en 2020, en médecine de ville, le taux de pénétration de ces médicaments n'est que de 23 %, bien loin de l'objectif de 80 % que le Gouvernement souhaitait atteindre d'ici 2022. Le présent amendement prévoit donc que la liste des biosimilaires substituables par les pharmaciens soit identique à celle des biosimilaires substituables par les médecins prescripteurs. Cette création logique d'un binôme prescripteurs-pharmaciens pour un suivi coordonné ne peut qu'améliorer l'accompagnement

Merci

dans la lignée de mon amendement précédent. Il est nécessaire de lever les freins potentiels, afin de permettre une mise en oeuvre rapide, effective et ambitieuse de ce dispositif. Le présent amendement vise donc à fixer par arrêté un échéancier précis, sur une période de deux ans, pour faire évoluer la liste des groupes biologiques similaires substituables, sur recommandation de l'ANSM. Cela permettra de tirer le plein potentiel de cette mesure, et d'apporter la lisibilité et la prévisibilité nécessaires aux acteurs, professionnels de santé et patients. L'application de ces mesures assurera ainsi le développement rapide de la pénétration des médicaments biosimilaires sur le marché de ville, en cohérence avec les objectifs déterminés par la stratégie nationale de santé.

Eu égard à son importance, à son impact sur la santé des patients et les parcours de soins, cet avis devrait être encadré dans son contenu comme dans ses modalités de publication. Il est ainsi essentiel que l'avis rendu par l'ANSM soit pris après consultation des associations de patients concernées. Les critères retenus par l'ANSM pour déterminer les groupes biologiques substituables doivent être publics, afin de pouvoir être connus des patients, de façon à garantir leur confiance comme la transparence des arbitrages rendus.

Je tiens à témoigner devant vous de l'importance de la transparence et de la pédagogie dans la substitution des médicaments. Il en avait été de même au moment du développement des médicaments génériques.

Il y a encore un vrai effort de promotion, d'explication et de pédagogie à faire tant auprès des médecins que des pharmaciens et des patients.

: La parole est à M. Olivier Henno. Cette disposition autorise la substitution par le pharmacien en initiation de traitement d'un médicament biologique par son biosimilaire. Cette substitution n'est possible que lorsque le prescripteur n'en a pas exclu la possibilité, mais le patient doit également pouvoir s'y opposer. Par ailleurs, la possibilité de substitution ne doit pas être ouverte dans le cas de pathologies lourdes et ne doit pas concerner les substances actives prévues dans le cadre de l'avenant 9 à la convention médicale parue au du 25 septembre 2021. À ce jour, cela concerne les six substances actives suivantes : étanercept, adalimumab, follitropine alfa, énoxaparine, tériparatide et insuline asparte.

J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ! Moi, quand je vais chez le médecin, ce n'est pas pour rédiger l'ordonnance ! Si le médecin me prescrit un produit et que le pharmacien me propose

Les enjeux sont importants et les travaux sur ce sujet doivent s'inscrire dans un climat de confiance. Les médicaments biosimilaires sont non pas identiques, mais équivalents aux médicaments biologiques de référence ; les changements de traitement ne sont donc pas sans conséquence pour les personnes malades.

à Mme Émilienne Poumirol. Cet article prévoit de valoriser les relocalisations en France et en Europe par des prix plus élevés pour les produits de santé issus des industries concernées.

Plusieurs points méritent d'être abordés. Tout d'abord, il nous semble fortement dommageable que l'assurance maladie, dont le déficit est toujours considérable et promis à le rester, soit ainsi mise à contribution

Elle sanctuarise donc inutilement une mesure qui a été pensée dans l'urgence de la crise sanitaire, en réponse aux nombreux dysfonctionnements des chaînes d'approvisionnement de médicaments essentiels provoqués par la hausse de la demande mondiale.

Vous l'aurez compris, nous sommes donc défavorables à la suppression de cet article ; il s'agit maintenant d'en examiner la rédaction. Quel est l'avis

Cet amendement vise à rendre publics les investissements en recherche et développement réalisés par l'État et à les prendre en compte- il s'agit d'une demande récurrente -dans la définition du prix des médicaments. La course au vaccin contre la covid-19 a révélé avec une ampleur sans précédent le rôle joué depuis toujours par la puissance publique dans le financement de la recherche et développement en santé. L'État contribue en effet très largement, de manière directe ou indirecte, au développement des médicaments mis sur le marché, par le le financement d'un système d'enseignement supérieur d'excellence formant des scientifiques et des chercheurs, par l'octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d'impôt recherche, par son investissement propre dans la recherche publique, par le partage des découvertes scientifiques, par le remboursement des produits de santé par la sécurité sociale. Ces sommes considérables investies par l'État ne sont pas rendues publiques ni prises en compte dans la négociation des prix des produits de santé avec les entreprises pharmaceutiques ; lesdits produits, faute d'une négociation éclairée,

Il faut arriver à mieux corréler le prix des médicaments à leur coût réel de recherche et de production. Or, aujourd'hui, de tels paramètres n'entrent pas en ligne de compte dans la fixation des prix et dans les décisions de remboursement prises par le CEPS.

prévoit déjà la transmission et la publication du montant des investissements dont ont bénéficié les entreprises. Avis défavorable sur ces deux amendements. Quel est l'avis